Émilienne Poumirol, Mme Angèle Préville, M. Claude Raynal, M. Christian Redon-Sarrazy, M. Lucien Stanzione, M. Jean-Claude Tissot, M. Jean-Marc Todeschini, M. Mickaël Vallet et M. Yannick Vaugrenard.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le début de la discussion des amendements sur ce projet de loi de finances m'incite à faire un point devant vous sur l'application des dispositions relatives à leur recevabilité financière et organique. La première partie du projet de loi de finances pour 2022 a fait l'objet du dépôt de 783 amendements au stade de la séance publique soit très peu, ont été déclarés irrecevables en application de l'article 40 de la Constitution, car ils étaient susceptibles de créer ou d'aggraver une charge publique

L'analyse de la recevabilité organique des amendements repose sur plusieurs critères. J'apprécie, en premier lieu, si l'amendement relève du domaine des lois de finances, tel qu'il est défini par l'article 34 de la LOLF, qu'il s'agisse d'un dispositif dispositif d'alignement de règles comptables, de la mise en oeuvre de nouvelles règles de facturation ou d'une demande de rapport ; 18 amendements ont ainsi été jugés étrangers au domaine des lois de finances. J'évalue ensuite si l'amendement est correctement placé et respecte la règle de bipartition. Aux termes de celle-ci, seuls les dispositifs fiscaux ayant une incidence sur les recettes de l'État en 2022 peuvent figurer en première partie.

principalement des collectivités territoriales ; 13 amendements ayant trait à un crédit d'impôt pour lequel le fait générateur n'intervient qu'à partir de 2022, et le remboursement de ce crédit auprès du bénéficiaire en 2023 5 amendements dont l'objet est la publication d'un rapport portant sur des dépenses, et non sur des recettes ; 20 amendements dont l'impact sur les recettes de l'État en 2022 est jugé nul pour d'autres motifs.

Inspiré par l'oeuvre politique de l'ancien président du Conseil Joseph Caillaux, il vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu (IR), à un taux faible, afin d'en élargir l'assiette. Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'IR, alors que celui-ci devrait rester l'impôt citoyen par excellence. 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable- inférieur à 6 311 euros annuels -peuvent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté, et de retisser les liens entre l'État et les citoyens. Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel,

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2021. Elle devrait être relativement neutre du point de vue budgétaire. Par ailleurs, les seuils de ces tranches sont revalorisés de manière à évoluer comme l'indice des prix hors tabac en 2021 soit de 1,4 %, ce qui neutralise les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.

Nous sommes convaincus du contraire ! D'où cette proposition d'augmentation du nombre de tranches, qui permet de solliciter les plus hauts revenus. Par exemple, sur 1 085 milliards d'euros de revenus déclarés, seuls 70 milliards sont prélevés au titre de l'IR. Nous sommes loin de la confiscation dénoncée régulièrement par les uns et les autres

Les socialistes du Sénat ont déterminé une courbe d'imposition permettant de sortir de l'imposition le quatrième décile de la population et de réduire l'imposition de manière dégressive pour les déciles 5 à 9, tout en augmentant de 1,9 milliard d'euros les recettes de l'État issues Cette proposition de rééquilibrage de l'imposition sur le revenu se traduit par une baisse d'imposition pour 14,8 millions de contribuables, en particulier ceux des classes moyennes. Il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays. Cet amendement tend à favoriser une redistribution saine et à renforcer le pouvoir d'achat de la quasi-totalité des Français, ce qui est bien légitime par les temps qui courent. Je compte donc, mes

Il apparaît ainsi légitime que les plus aisés contribuent un petit peu plus à la solidarité nationale. Cet effort demeure, au surplus, relativement minime. Redistribution, encore et toujours ! Quel est

Le scrutin est clos.

de défendre un contre-projet qui se veut féministe. Le principe en est simple : faire en sorte que notre système fiscal, au lieu de graver dans le marbre, voire d'aggraver, les inégalités de genre, les résorbe et les corrige. Il est possible de défiscaliser une aide alimentaire quand on la paie, mais, bizarrement, elle est considérée comme un revenu quand elle est reçue. Or le dernier rapport sur les ruptures familiales du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) établit que, dans 97 % des cas, la pension alimentaire est versée par les pères. C'est donc la double peine : en plus de devoir mener de front vies familiale et professionnelle, recevoir une pension alimentaire pour la garde des enfants signifie payer plus d'impôts sur le revenu. À l'inverse, ne pas avoir la garde des enfants permet de se focaliser entièrement sur sa vie professionnelle, avec en prime un abattement fiscal ! Je

stables. Notre système fiscal aggrave certaines inégalités, et il est temps que cela cesse. Cet amendement vise donc à ce que le bénéfice d'une pension alimentaire ne soit plus comptabilisé dans le calcul de l'impôt sur le revenu et que, à l'opposé, le paiement d'une pension alimentaire le soit.

est un mécanisme dont le caractère vertueux a fait ses preuves. Il peut également s'avérer un outil de relance particulièrement performant. Force est de constater qu'au vu du prix moyen d'un déjeuner, soit 14 ou 15 euros, de l'augmentation des prix dans l'alimentation et du contexte économique, il convient de rehausser la valeur maximale du titre-restaurant. Le présent amendement a ainsi pour objet de rehausser le montant maximum de la participation patronale aux titres-restaurants à 7,50 euros, au lieu de 5,55 euros. Cette mesure permettrait de revaloriser le pouvoir d'achat des salariés, tout en apportant aux secteurs de la restauration et de l'alimentation un soutien efficace à leur activité.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les pensions versées sont soumises à une contribution, à la charge du bénéficiaire, de 7 % pour les rentes comprises entre 500 et 1 000 euros par mois, de 14 % pour celles comprises entre 1 000 et 24 000 euros par mois, et de 21 % au-delà de 24 000 euros. Ce mécanisme visait à l'origine à taxer les retraites chapeaux, mais il apparaît injuste pour les retraites plus modestes, alors que les retraites de la fonction publique ne sont pas concernées. En outre, outre, il s'est appliqué aux retraites en cours. Il concerne environ 200 000 retraités, dont le revenu de remplacement a été lourdement touché. Si le présent amendement ne propose pas de supprimer ces contributions de 7 % et 14 %, il vise néanmoins à les rendre déductibles de l'impôt sur le revenu des ménages. Il nous semble qu'il s'agit d'une mesure de justice fiscale, face à une situation pénalisante pour nombre de nos concitoyens.

ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont la quasi-totalité des revenus est de source française, et qui ne bénéficient pas de mécanismes de nature à réduire leur imposition dans leur État de résidence, d'être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Ils peuvent ainsi bénéficier de réductions et de crédits d'impôt, contrairement au reste des non-résidents fiscaux. Le critère de la domiciliation crée forcément des inégalités fiscales entre catégories de non-résidents.

À ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce, généralement liées au versement d'une pension alimentaire, ne sont pas déductibles des revenus soumis à l'impôt.

réciprocité n'est pas possible entre la France et un pays tiers. Autrement dit, un Français résidant dans un autre pays ne bénéficie pas des mêmes avantages. L'amendement n°

à domicile, les personnes âgées en situation de perte d'autonomie peuvent quant à elles bénéficier d'un crédit d'impôt depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d'autonomie demeurant anciennement à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement, et ceci en raison d'un accident de la vie ou de l'apparition de troubles du comportement sévères. Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de réduction d'impôt en crédit d'impôt pour les personnes âgées en perte d'autonomie hébergées en établissement. Il s'agit ici d'assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l'entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

dans les établissements d'hébergement médico-sociaux.

Bilhac. Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par notre collègue Éric Gold en début d'année, malheureusement rejetée par le Sénat il y a quelques semaines, qui visaient à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et de loisirs dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Vous le savez, avec la crise sanitaire, de nombreuses associations ont vu leurs adhésions non renouvelées, et connaissent des difficultés financières.

et en France, afin de préserver une équité fiscale entre résidents et non-résidents. cet amendement correspond à l'article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020.

de France. Dans une période de crise, il n'y a pas de bonne raison de ne pas encourager la générosité des redevables français, où qu'ils se trouvent.

soient exclus. La doctrine fiscale prévoit que les bénévoles puissent bénéficier d'un défraiement de leurs déplacements dans le cadre d'activités associatives, sur présentation de justificatifs fournis par lesdites associations. face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 avait étendu le champ de l'article L. 3131-10 du code de la santé publique, relatif à la réserve sanitaire, aux professionnels de santé bénévoles. Il est ainsi question d'actualiser pertinemment les dispositifs relatifs à l'action des bénévoles. Pour reconnaître leur rôle dans la campagne de vaccination, le présent amendement prévoit d'étendre à leurs frais de déplacement le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons aux associations prévue à l'article 200 du code général des impôts. Les détails de l'application de cette mesure seraient quant à eux renvoyés à un décret.

La suppression du crédit d'impôt pourrait conduire les personnes les plus fragiles à solliciter les caisses afin de bénéficier d'aides financières sous condition de ressources et de critères donc important de prendre en compte ces demandes tout à fait légitimes, en signe de solidarité. Les services aux personnes sont très importants.

le travail et la vie privée, tout en luttant contre l'économie souterraine. Au fur et à mesure, le bénéfice de cette dépense fiscale a été étendu aux personnes en recherche d'emploi puis aux retraités.

élever seul ses enfants signifie un risque accru de précarité, notamment quand on est une femme : 45 % des enfants vivant avec leur mère sont sous le seuil de pauvreté, ce qui est également le cas de 22 % de ceux

des études ou avoir un peu de temps pour eux. C'est pourquoi cet amendement de ma collègue Mélanie Vogel vise à faire passer de 50 % à 80 % le taux du crédit d'impôt relatif aux services à la personne pour les familles monoparentales.

pour les dépenses assumées par les personnes seules avec un enfant, me paraît relativement inadapté. Je ne suis personnellement pas favorable à ce que l'on attribue plusieurs finalités

à un même taux et sur une même assiette. Évitons de rendre le dispositif peu lisible, pour ne pas dire plus

et permettre cette insertion sur l'ensemble du territoire français, dans le contexte de réduction du budget alloué au sport. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans leur convention de mécénat relative à l'accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, dont plus de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté.

Ce frein pénalise en particulier les sportifs peu ou non connus du grand public, qui représentent l'avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s'inscrire dans une démarche de parrainage commercial. À ce jour, l'état du droit ne donne pas au mécène la possibilité d'associer le nom d'un sportif identifié à son action de mécénat. Cet amendement, dû à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Lozach, a donc pour objet de conforter la possibilité offerte à un mécène d'affecter son don à un sportif de haut niveau en particulier,

de plus en plus pressantes à mesure qu'approche la campagne présidentielle, toutes les pistes semblent bonnes à prendre pour améliorer l'ordinaire des salariés. La défiscalisation et la « désocialisation » des pourboires en sont la dernière illustration

la pratique du pourboire est fortement préjudiciable, en ce qu'elle « désocialise » le salaire fixe qui doit être garanti à tout employé. Cette annonce a été faite par le Président de la République lors du Salon international de la restauration et l'hôtellerie, le but étant d'accroître le pouvoir d'achat des salariés afin de contribuer à attirer des candidats qui font cruellement défaut, le rappelle, près de 110 000 postes ne sont toujours pas pourvus dans ce secteur sous tension. Toutefois, la mesure proposée est inique, puisque l'on constate que la pratique du pourboire s'essouffle, surtout depuis que le service a été inclus dans la note, en 1987, et que le pourboire est devenu totalement optionnel. En conclusion, c'est sur les conditions de travail et de rémunération qu'il faut s'interroger, afin de remédier au manque de personnel dans les secteurs en tension, et ce n'est pas l'artefact proposé dans cet article qui changera fondamentalement l'attractivité de ces métiers.

la défiscalisation des pourboires risquerait d'accroître la précarité des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration, puisque le bénéfice de la mesure serait réservé aux travailleurs percevant moins de 1,6 ; on peut donc imaginer que la stratégie des employeurs consiste, pendant les deux prochaines années, à fixer systématiquement le montant des salaires juste au-dessous de cette limite.

La réalité, nous la connaissons tous : les paiements en numéraire sont en voie d'extinction ou, en tout cas, décroissent de manière extrêmement forte et la période d'épidémie que nous avons vécue a accéléré les paiements par voie électronique, notamment par carte bancaire pose un problème d'attractivité pour les professions qui peuvent bénéficier de pourboires, puisque ceux-ci pouvaient représenter des revenus additionnels assez importants et que le paiement par carte bleue n'incite pas au versement d'un pourboire.

monsieur le ministre, je constate que, aujourd'hui encore, 50 % des transactions commerciales se font en espèces.

Cet amendement vise à étendre l'avantage fiscal aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d'une attestation établissant que leurs époux pouvaient prétendre à la qualité de combattant de leur vivant.

ans. La loi de finances pour 2020 avait déjà permis aux conjoints survivants d'anciens combattants décédés entre 65 et 74 ans de bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Nous proposons d'étendre ce dispositif aux conjoints d'anciens combattants décédés avant l'âge de 65 ans, mais toujours

I-238 rectifié, plus restreint, tend à ouvrir la demi-part fiscale à tout conjoint survivant pouvant établir que le conjoint décédé aurait pu prétendre à la qualité de combattant.

conduisait « à créer dans certains secteurs, notamment le commerce et l'artisanat, une concurrence déloyale avec les professionnels qui sont soumis à des règles sociales, fiscales, et des normes différentes de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), Alain Griset, ajoutait encore que ce régime « permet, sans véritable contrainte, de légaliser le travail dissimulé et procure des avantages particuliers

afin d'en faire un tremplin pour le démarrage d'activité et la création d'entreprise, mais pas plus. Quel

M. Emmanuel Capus. L'article 4 vise à allonger les délais au cours desquels les travailleurs indépendants en microentreprise peuvent choisir entre un régime d'imposition micro ou réel-

par souci de cohérence et de simplification. Le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d'une SCOP est prévu aux articles 160 et 210 D du code général des impôts. L'article 160 précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée, pour l'associé qui se retire de la société à l'issue de sa transformation en SCOP, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. L'article 210 D, quant à lui, applique à l'écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps, calquée sur le régime des fusions. L'Autorité des normes comptables a récemment publié un règlement appliquant aux SCIC le même régime qu'aux SCOP. Dans le même esprit, nous souhaitons simplifier l'ensemble du dispositif en harmonisant les régimes fiscaux applicables aux associés des deux

Or le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d'une SCOP inclut également les articles 160 et 210 D du CGI, qui précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais qui n'ont pas d'effet sur la base ou le taux d'imposition en ce qu'ils ne renvoient pas à la loi du 10 septembre 1947.

les SCIC peuvent être détenues par des personnes morales, en particulier des entreprises. La neutralisation des plus-values réalisées lors de la création n'est, de ce point de vue, pas forcément souhaitable.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés. Un dispositif de déduction de l'impôt sur les sociétés des intérêts d'emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding.

Capus. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles les SCOP constituent leurs provisions pour investissement. En l'état actuel du droit, les montants qui y sont consacrés dépendent de ceux qui sont versés à la réserve de participation. Cet amendement tend à prendre pour base de calcul les sommes affectées à la réserve légale ou au fonds de développement. Le changement de base de calcul devrait permettre aux SCOP d'augmenter leurs provisions pour investissement et donc,, leurs capacités effectives d'investissement. Quel est l'avis de la commission

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa et de la déduction pour épargne, qui l'a remplacée en 2019, lesquelles permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique pour ne l'utiliser que dans des conditions prévues par la loi.

précédentes. Des modalités de versements, de contrôles et de sanction sont bien évidemment prévues. En basant leur dispositif sur les « sur-bénéfices » engrangés du fait de la crise, les auteurs de la proposition de loi saluent directement les actions menées par plusieurs entreprises d'assurance, dont les efforts viendront

et pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et à celui d'associations faisant oeuvre sociale, dont les services sont particulièrement demandés en cette période. doivent pouvoir compter sur l'engagement sans faille de l'État et des collectivités à leurs côtés. La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité.

Cet amendement vise à réorienter la comptabilité des entreprises afin de cesser de l'asseoir sur la seule vision actionnariale et de la centrer enfin sur la réalité économique.

Le choix de l'Union européenne, en 2002, de déléguer à l'IASB la définition des normes comptables des plus grandes entreprises européennes pose donc un double problème : de souveraineté, d'une part, et d'alignement sur la valeur actionnariale, d'autre part. part. La réévaluation des actifs ne fait en réalité que produire de la valeur fictive, inutile pour l'entreprise en tant que projet commun. Elle correspond à une interprétation très orientée de l'image fidèle, focalisée sur la valeur de marché et non sur la réalité du projet de l'entreprise

et comment il est utilisé pour l'activité de l'entreprise. Dans une vision centrée sur l'actionnaire, la comptabilité ne cherche qu'à montrer ce que possède l'actionnaire, selon une évaluation permanente par les marchés, sans aucun impact sur la réalité de l'activité de l'entreprise. Ainsi, le seul intérêt de la réévaluation des actifs est de créer de la valeur pour l'actionnaire. Cela ne sert ni la relance ni le soutien d'urgence à l'économie. Dans ce cadre, il est clair que la neutralisation du surcroît d'imposition est de nature à créer de nombreux effets d'aubaine. Si elles ne souhaitent pas être imposées, les entreprises n'ont qu'à s'abstenir de procéder à de telles réévaluations. Si l'on veut sincèrement décarboner l'économie, prendre en compte la destruction des services écosystémiques fournis par la nature et améliorer les conditions de travail et l'égalité femme-homme, il est essentiel que la comptabilité se détache du seul objectif actionnarial.

à l'ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu. Il vise donc à faciliter les fusions d'exploitations par la voie sociétaire des avantages fiscaux, ce qui semble favoriser la concentration du foncier agricole et l'agrandissement des fermes, allant ainsi à l'encontre des objectifs d'installation et de partage du foncier, qui doivent pourtant être le socle des politiques agricoles. Plutôt que de viser la concentration, nous pensons qu'il faut favoriser une situation dans laquelle les exploitations sont nombreuses, pour préserver l'emploi, l'environnement et la vitalité des territoires ruraux. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

parallèle un ensemble de technologies basées sur l'existence de capteurs permettant, avec des algorithmes qualifiés, de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d'agir buse par buse.

L'enveloppe initiale de 135 millions d'euros a bénéficié d'un abondement de 80 millions d'euros supplémentaires,

général des impôts prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation. Cela procure Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente. Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s'appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l'irrégularité des revenus agricoles. Or ces dispositifs ont une finalité totalement différente. Il s'agit, d'un côté, d'alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente, de l'autre, de pallier les conséquences d'une irrégularité des résultats, liée notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

de sa coopérative. En effet, quand les prix de l'année sont au-dessus d'un prix de référence, l'exploitant ne reçoit que le prix de référence, et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l'épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative. En cas de retrait de l'associé de sa coopérative ou lorsqu'il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l'exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l'intégralité du montant de la déduction afférente à l'épargne en créances, puisqu'il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction, donc réduire son résultat imposable, qu'à hauteur de 41 400 euros, une DEP classique, sur compte bancaire. La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement

alors même que l'exploitant n'a pas utilisé son épargne de précaution, ayant simplement été contraint légalement de la réintégrer. Par cet amendement, il s'agit donc de permettre à l'exploitant de transférer, notamment dans l'hypothèse d'un retrait, le montant des créances DEP qu'il détient sur sa coopérative sur le compte d'épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l'instar de ce que la loi prévoit pour l'épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers. L'amendement n° I-510 rectifié n'est pas défendu. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n°

qui doit être inscrite sur un compte bancaire. Pour les coopérateurs, il arrive que cette épargne soit constituée de créances détenues sur la coopérative. Lorsque les contrats

contreparties des déductions pour épargne de précaution. Le seul moyen de neutraliser cette conséquence est de pratiquer une nouvelle déduction, mais sous le régime limitatif prévu par l'article 73 du code général des impôts, en particulier un plafond annuel. Le dispositif de la DEP est déjà très souple d'utilisation et la créance détenue auprès d'une coopérative, qui peut être reprise par un exploitant agricole,

Le présent amendement vise à inciter à l'utilisation de l'épargne de précaution dans le cadre d'un aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, des aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l'offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds dédié aux calamités. Si la loi de finances pour 2019 a mis en oeuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution, l'expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants, dans la période de six à vingt-quatre mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d'inondation ou la survenance d'une maladie. Le dispositif vise ainsi à modifier les conséquences de l'utilisation de l'épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d'un aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, qui serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus.

Je précise en complément que la conjoncture n'a sans doute jamais été aussi propice au changement proposé, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l'évolution des mécanismes de soutien à venir.

d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. Il s'agit de défiscaliser ces sommes, puisqu'elles ne seraient pas réintégrées au résultat fiscal. La DEP

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à renforcer le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles. L'agriculture française est confrontée à l'enjeu crucial de renouvellement des générations et d'installation de paysans. Alors que le nombre d'exploitants baisse de 1 % à 3 % par an et qu'on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l'attractivité à la profession. Un crédit d'impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d'un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cette mesure a permis de développer l'accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Cet amendement vise à étendre cette mesure, par une prise en compte à 100 % des dépenses de remplacement pour les quatorze premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale. Les salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en effet un vivier de renouvellement des générations.

Dans la version actuelle du crédit d'impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d'agriculteurs, qui renoncent ainsi à prendre des congés. Or, on le sait, nombre d'agriculteurs souffrent de mal-être au travail, notamment du fait d'épuisement professionnel. Le rapport sénatorial de nos collègues Henri Cabanel et Françoise Férat de nos collègues Henri Cabanel et Françoise Férat souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Il estime ainsi qu'« une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d'un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de " souffler tout l'esprit de cet amendement, qui, face à une situation souvent difficile pour nombre d'exploitants agricoles, vise à renforcer l'accessibilité au remplacement pour congé. Son adoption permettra en outre de renforcer l'attractivité du métier d'agriculteur, à l'heure où la moitié des exploitants agricoles partira à la retraite dans les dix prochaines années. Il tend également, alors que ce crédit d'impôt doit prendre fin en 2022,

trois amendements. Ces amendements visent à définir des conditionnalités environnementales pour le crédit d'impôt prévu dans le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. L'amendement n° I-768 rectifié tend à conditionner ce dispositif à l'absence de coupes rases, car cette pratique conduit au remplacement d'un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que M. Labbé et les spécialistes savent que des itinéraires techniques d'amélioration à moindre impact sont possibles. Il tend également à le conditionner à des pratiques permettant de favoriser la diversification des peuplements, et donc la résilience des forêts au changement climatique. L'amendement n° I-767 rectifié prévoit une conditionnalité sur la question de la commercialisation, pour faire en sorte que les personnes s'engagent à commercialiser à un opérateur de transformation situé

objectifs d'Aichi et les engagements de la France au titre des accords de Paris. Elle s'inscrit dans l'esprit de la feuille de route du ministère de l'agriculture pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Ces amendements sont cohérents avec la stratégie de l'Union européenne pour les forêts, qui est en cours de discussion,

que le crédit d'impôt soit le bon outil fiscal pour soutenir les industries de transformation de bois de notre pays. Vous le savez,

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques ou aux coûts économiques et environnementaux d'une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative. Il existe bien des dispositifs d'exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton ou une commune limitrophe. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des propriétaires qui le recevra. appellation d'origine contrôlée (AOC) peut s'étendre sur des territoires dépassant la limite d'un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d'exonération ou n'ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

La limitation cantonale répond, vous le savez, à des problématiques strictement administratives. Certes, les cantons ont évolué sous l'effet des réformes. En l'occurrence, la taxe de publicité foncière, qui constitue un droit de mutation, est versée aux départements

cette aide doit s'appliquer le plus tôt possible, dès 2022, l'agriculture biologique ayant subi, les années précédentes, la fin du financement national de l'aide au maintien. De plus, l'agriculture biologique sera moins soutenue, dans la version actuelle du plan national stratégique, agricole commune (PAC). Il convient donc de sécuriser le crédit d'impôt pour toute la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu'en 2027. Enfin, le montant de 5 000 euros paraît plus justifié au regard de la fin de l'aide au maintien et des atouts de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est un outil reconnu de la transition agroécologique, comme l'a rappelé le dernier rapport de France Stratégie sur sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie, qui affirme l'efficacité de l'agriculture biologique, définie comme « la plus performante d'un point de vue économique et environnemental aujourd'hui ». Ce crédit d'impôt se justifie ainsi largement par les nombreuses externalités positives associées à l'agriculture biologique, qu'il s'agisse de la qualité de l'eau, de la protection des pollinisateurs, de la préservation des sols, la réduction des pollutions de l'air ou de la qualité de l'alimentation. Enfin, le Pacte vert pour l'Europe fixe un objectif pour 2030 de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique : il est donc important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et en augmentant le crédit d'impôt bio.

nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition et exclut, de fait, les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d'imposition sur les sociétés. Or ces entreprises sont tout aussi sujettes aux divers aléas climatiques et économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face. Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l'imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l'imposition sur les sociétés d'utiliser le dispositif d'épargne de précaution est en contradiction avec l'incitation des pouvoirs publics. Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d'affaires global de la société. La

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d'affaires global de la société.

les autres héritiers s'engagent à conserver les biens transmis en les laissant à la disposition des repreneurs pendant une longue durée, soit dix-huit ans au moins. La fiscalité qui s'applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène. En effet, les biens loués par bail à long terme bénéficient d'une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d'une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans. Le présent amendement vise à prévoir un engagement beaucoup plus long d'au moins dix-huit ans, ce qui constitue une garantie pérenne de stabilité pour l'exploitation familiale, en contrepartie d'une exonération totale des droits de mutation.

La stabilité du foncier attaché aux exploitations est indispensable à la pérennité de celles-ci. Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s'engagent à les conserver plus longtemps. Actuellement, l'exonération de 75 % s'applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d'appliquer l'exonération de 75 % jusqu'au double de ce plafond, soit 600 000 euros lorsque les bénéficiaires s'engagent à doubler la période de conservation, c'est-à-dire dix ans au lieu de cinq ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l'engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l'ayant cause.

à 600 000 euros l'exonération de 75 % sous la condition d'une durée de conservation minimale portée de cinq à dix ans. Les conditions de transmission ont été améliorées par la loi de finances pour 2019, avec une revalorisation substantielle du plafond de la déduction à 75 %. Elles sont d'ailleurs plus avantageuses dans le champ agricole que pour d'autres secteurs puisque l'engagement de conservation est moins exigeant que l'engagement d'exploitation généralement posé. ce type de mesures qui conditionnent un avantage fiscal à des durées de conservation peut se retourner contre les bénéficiaires,

apprécier ces exonérations à l'aune des engagements personnels du bénéficiaire, la simple conservation des biens n'étant pas équivalente à un engagement d'exploitation personnelle. Dans un devoir de vigilance, j'en sollicite le retrait. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu'elle débouche sur une imposition partielle et que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement. Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l'addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l'impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre. La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L'achat par l'exploitant, lorsqu'il est possible, absorbe une grande partie, voire la totalité des capacités financières de l'entreprise, et obère son développement. L'achat par d'autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

haute valeur environnementale (HVE), introduit dans le PLF pour 2021. En effet, cette certification n'a pas fait ses preuves et de nombreux travaux parus au cours de l'année 2021 confirment sa faible performance,

Choisir. Tous ces rapports démontrent que les effets du label HVE sont très faibles, voire inexistants, et peu avérés. Il peut être intéressant de valoriser et d'encourager des pratiques intermédiaires entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, ce qui est l'objectif affiché de la HVE. Mais le cahier des charges de cette certification tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas la garantie d'un véritable progrès. La réforme du cahier des charges engagée par le Gouvernement ne donne pour l'instant aucune garantie et interviendra trop tard pour que le crédit d'impôt ait une réelle efficacité. La somme accordée à ce crédit d'impôt pourrait financer des dispositifs plus cohérents et plus performants ; c'est pourquoi nous en demandons la suppression.

: La parole est à Mme Sylvie Vermeillet. Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd'hui grandement fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel. Cet amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment les entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir.

Ce mécanisme, en permettant une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers, notamment du financement de programmes d'investissement. Un dispositif similaire existe en Allemagne et en Autriche, et concourt, avec d'autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française. Quel est l'avis de la commission

dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros. La provision proposée pourrait être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal.

Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d'une alimentation saine et durable. Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle,

et du travail (Anses) pour permettre la mise en oeuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l'agent comptable de l'Anses. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an. La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1 janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques, la DGFiP. Il n'était en effet pas opportun que l'Anses, chargée d'évaluer et d'autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure doit également permettre de contribuer à l'efficience du recouvrement et du contrôle de l'assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité. Pour autant, les frais de recouvrement prélevés par la DGFiP ne seraient pas cohérents avec la réalité des coûts induits par cette activité. général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l'État. de recettes engendrée serait ainsi de 0,5 million d'euros par an pour le fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques et de 0,2 million d'euros par an pour la phytopharmacovigilance. C'est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5

le taux réduit est déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale. Un taux de recouvrement plus important diminuerait les montants consacrés à la phytopharmacovigilance, ainsi qu'au fonds d'indemnisation.

n° I-423 rectifié . Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s'acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l'article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l'évaluation et de l'autorisation de ces médicaments par l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), qui relève de l'Anses. Le barème des taxes n'a pas été réévalué depuis 2013 et ne couvre désormais plus les coûts de cette activité. Par ailleurs, il est inutilement complexe. Le règlement (UE) 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier prochain, procède à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif. mesure d'adaptation et de simplification du barème des taxes applicables aux médicaments vétérinaires apparaît indispensable. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais avec une entrée en vigueur différée.

devons lutter contre la concentration du CIR par les grandes entreprises, car la recherche et l'innovation sont pour elles un élément de compétitivité prépondérant. La recherche sert à gagner des parts de marché et à réaliser des gains de productivité ; c'est un phénomène économique. L'argent public doit non pas se substituer à l'investissement privé, mais l'encourager pour orienter les décisions d'investissement vers des activités socialement et écologiquement justes.

émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

du CIR : « Dans le contexte de la planification d'après la guerre mondiale, l'État a joué un rôle structurant en finançant massivement et de façon extrêmement sélective certaines filières industrielles- nucléaire, aéronautique, informatique et communication,

d'impact significatif sur la valeur ajoutée et l'investissement ». L'innovation se fait souvent en dépit de toute logique environnementale et climatique. Les dépenses de recherche doivent être vertueuses. C'est pourquoi cet amendement vise à appliquer une conditionnalité au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche en excluant certaines activités en lien avec la production et la consommation d'énergie fossile. Cette exclusion permettra de retirer les dépenses de recherche et de développement d'une entreprise si celles-ci sont incluses dans une activité pouvant être facilement caractérisée. Elle Elle empêchera aussi de soutenir, par le crédit d'impôt, les dépenses de recherche et de développement de ce secteur dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

et 2015, 8 868 entreprises ont bénéficié au moins une fois de ce dispositif, pour un montant total d'exonérations de cotisations sociales patronales de 1,5 milliard d'euros. Pour la seule année 2015, quelque 3 487 entreprises se sont réparti 160 millions d'euros d'exonérations au titre des dépenses de personnel. Si 55 % des entreprises atteignent l'âge limite du dispositif, elles ne sont que 25

innovante aux entreprises de plus de 250 salariés. Je rappelle que, aujourd'hui, 90 % des jeunes entreprises innovantes emploient moins de 20 salariés.

Le présent amendement vise à réguler le régime des sociétés mère-fille, source particulière de l'érosion des bases imposables en matière d'impôt sur les sociétés pour les groupes disposant de filiales hors de l'Union européenne. Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20,2 milliards d'euros. À titre de comparaison, le produit de l'impôt sur les sociétés est évalué en loi de règlement à 33,5 milliards La dépense fiscale concernée représente donc 60,3 % de l'ensemble de l'imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le dispositif proposé consiste à limiter l'actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l'Union européenne, à rétablir, pour les pays hors de l'Union et les flux concernés, un mécanisme de crédit d'impôt, lequel limitera les déductions fiscales, et, enfin, à plafonner ce crédit d'impôt. Ainsi organisé, l'amendement respecte le droit de l'Union européenne et sa pertinence, pour ne pas dire sa nécessité, laquelle ne fait aucun doute.

l'accord trouvé au sein de l'OCDE sur les règles du pilier 2 doit permettre de réduire l'efficacité des pratiques de transfert de bénéfices, auxquelles les amendements en discussion entendent s'attaquer.